Mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque, qui doit couvrir le nez, est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs s'exprimant à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents réunie le 1 décembre dernier.

? ». Je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé d'expérimenter une proposition du groupe de travail sur la modernisation des méthodes de travail du Sénat. En application de cette proposition, le groupe CRCE disposera d'un temps de présentation de huit minutes. le Gouvernement aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l'auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répliquer pendant une minute. Le temps de réponse du Gouvernement à l'issue du débat est limité à huit minutes. Le groupe auteur de la demande de débat disposera de cinq minutes pour le conclure.

se traduit par une dégradation des conditions de travail, par une mise sous tension des services publics, notamment à l'hôpital, et par la multiplication des plans de licenciements. Je pense notamment aux anciens salariés de France Loisirs, dont 118 du site de Noyelles-sous-Lens, dans mon département du Pas-de-Calais, qui ont été licenciés. Et avec quel cynisme : un courrier reçu le 24 décembre au matin et l'accusé de réception le 31 ! Joyeux Noël et bonne année à tous ces salariés ! Je pense également aux métallos de la Société aveyronnaise de métallurgie (SAM), qui employait 350 personnes dans l'ancien bassin minier de Decazeville. Ils ont passé le réveillon du nouvel an dans leur usine, usine, occupée depuis fin novembre à la suite de la liquidation de cette entreprise sous-traitante de Renault, qui a pourtant bénéficié de 5 milliards d'euros d'aides de l'État. Je pense enfin aux salariés des sites Arkema qui, en grève depuis le 16 décembre,

La liste est longue et je m'arrêterai là. La pandémie de covid-19 a entraîné un renforcement des inégalités entre les salariés, qui ont subi une dégradation de leurs conditions de vie, et les entreprises du CAC 40, qui ont réalisé, au premier semestre 2021, 60 milliards d'euros de profits. Ces mêmes entreprises qui ont bénéficié d'aides publiques ont pourtant licencié 60 000 salariés dans le monde, dont 15 000 en France. Face à l'accumulation des richesses entre les mains d'un petit nombre et à la dégradation des conditions de vie du plus grand nombre se pose la question d'un meilleur partage des richesses et du travail. La durée de travail est au coeur des luttes de classes ; pourtant, la crise sanitaire semble donner un sens nouveau à l'aspiration à la réduction du temps de travail. la généralisation du recours au télétravail a entraîné un affaiblissement des frontières entre vie personnelle et vie professionnelle, mais a également favorisé l'expérience d'une réduction du temps de travail au profit de la vie familiale. Certaines entreprises ont compris l'intérêt d'améliorer le bien-être de leurs salariés. La société d'agencement en bois Design Bois s'est ainsi créée en 2006 sur le concept de la semaine de quatre jours.

Ainsi un quotidien économique titrait-il, le 10 décembre dernier : « Ces entreprises qui testent la semaine de quatre jours ». Je vous donne lecture du chapeau : « Discrètement, depuis la pandémie, de plus en plus de PME testent la suppression du vendredi ou d'un jour de travail dans la semaine. Les patrons qui l'ont mise en place revendiquent plus de bien-être et plus d'efficacité chez leurs salariés. C'est aussi un argument dans la guerre actuelle des recrutements. » Le journal rejoint ainsi la campagne menée par la Confédération générale du travail (CGT) en faveur de l'abaissement du temps de travail. Pour la CGT, la réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire permettrait à toutes et à tous de travailler. En France, le nombre annuel d'heures supplémentaires est estimé à 800 millions, soit 500 000 équivalents temps plein. En réduisant le temps de travail, on permet des créations d'emplois, on favorise l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l'égalité dans l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, et on permet aux salariés de disposer des temps nécessaires pour s'investir sous différentes formes dans la vie sociale. Cette campagne syndicale rejoint notre projet politique de transformation sociale de la société. Nous avons conscience des résistances qui existent du côté du patronat, relayées par le Président de la République : les Françaises et les Français, selon eux, travailleraient moins que leurs voisins. Cette affirmation est fausse, comme le démontrent les statistiques d'Eurostat, qui mesure le temps de travail à 37,4 heures en France, contre 37,3 en Espagne, 37 en Italie et en Belgique, 35 en Allemagne et 30,4 aux Pays-Bas. Il est donc non seulement faux de dire que nous travaillons moins, mais c'est même l'inverse ! La réduction du temps de travail n'est ni l'ennemie du salaire ni celle de l'emploi. Contrairement à ce que certains candidats à l'élection présidentielle peuvent affirmer, peuvent affirmer, elle n'obère pas l'augmentation des salaires, au contraire. Il suffit de regarder les chiffres de l'Insee pour s'en convaincre. Le passage aux 35 heures a entraîné un gain de productivité de 4 % à 5 % pour les entreprises, plaçant la France au deuxième rang mondial pour la productivité horaire, devant les États-Unis et l'Allemagne. Les 35 heures ont permis un fort développement de l'économie de la culture, des loisirs et du tourisme grâce au temps libre dégagé, ainsi que la création de 350 000 et 500 000 équivalents temps plein travaillé. La réduction du temps de travail ne doit pas se traduire par une hausse de l'intensification du travail, bien au contraire. C'est en libérant la parole des salariés sur leur travail, en leur donnant de nouveaux droits d'intervention, que l'on contribuera à éviter les dérives de la mise en place des 35 heures, par exemple dans les secteurs des services et de l'industrie ou à l'hôpital public. La réduction du temps de travail est plus que jamais à l'ordre du jour. Pendant la crise sanitaire, elle a constitué, sous forme de chômage partiel, la mesure principale de gestion de l'emploi, avec le télétravail ou le travail à domicile. Ainsi les données de l'Insee montrent-elles que, lors du premier confinement, de mi-mars à mi-mai 2020, le nombre d'heures travaillées par personne a diminué d'un tiers,

d'une vie sociale, culturelle, sportive et démocratique. Diminuer le temps de travail, c'est améliorer les conditions de vie de chacune et de chacun en créant massivement des emplois à temps plein, bien rémunérés, plutôt que des contrats à temps partiel extrêmement précaires. En réduisant le temps de travail de chacun, on favorise une meilleure répartition du travail disponible et on crée les conditions permettant d'atteindre un réel plein emploi.

À quoi bon faire travailler les gens plus longtemps quand tant de jeunes attendent un emploi ? Partager le travail et les richesses constitue un enjeu fondamental pour l'épanouissement de l'humanité. Dans la suite

le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vais vous donner lecture de l'intervention de mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, empêché ce jour, mais dont je partage la brillante analyse. Le partage du travail : un outil pour le plein emploi ? C'est une question légitime que l'on doit se poser, mais ledit partage est-il bien la bonne réponse pour atteindre le plein emploi aujourd'hui ? Premier constat : le temps de travail a diminué de moitié en cent soixante-dix ans grâce à l'action syndicale et à celle des pouvoirs publics. De 3 021 heures en 1851,

de ces lois a sauvé des emplois. La seconde en a créé 100 000, 200 000, 300 000- les experts ne se sont jamais mis d'accord. Mais elle a sûrement handicapé certains secteurs face à la concurrence étrangère, en augmentant le coût du travail. Deuxième constat : en 1995, dans un rapport du Commissariat général au plan rédigé par le journaliste Jean Boissonnat, il était précisé, entre autres, que le mouvement séculaire de réduction du temps de travail se poursuivrait plutôt sous la forme de temps variables et choisis. Vingt-cinq ans plus tard, cela reste d'actualité. Mais Jean Boissonnat soulignait également que l'erreur de tous ceux qui voulaient partager le temps de travail était de considérer celui-ci comme un gâteau de taille constante, alors que le meilleur moyen d'augmenter le nombre de parts est d'augmenter la taille du gâteau. Aucun doute, c'est la croissance qui permettra le plus sûrement de créer des emplois. Troisième constat : certains doutaient, voilà peu, du retour à la croissance. Or la croissance est là, plus forte qu'espérée, +6,7 % en 2021.

La question à se poser est donc tout autre : ne faut-il pas repenser le travail, le réorganiser, dans ces secteurs qui manquent d'attractivité ? Certains, sans attendre, quand c'est possible, modifient les horaires et les conditions de travail, augmentent la rémunération. Faut-il d'ailleurs appeler « travail » la seule activité donnant lieu à rémunération ? Selon la vision de l'économiste et ingénieur Marc de Basquiat, l'activité, qui prend de multiples formes, doit être systématiquement valorisée un revenu universel de base ; mais c'est là un autre débat.

Quant au partage des richesses et des responsabilités dans l'entreprise, c'est-à-dire la participation et l'intéressement, il est à nouveau d'actualité ; je m'en réjouis. Il faut que chaque homme ou femme « trouve sa place dans la société, sa part et sa dignité », comme disait le général de Gaulle.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, notre pays, au fil de son histoire, s'est honoré de toutes les avancées sociales liées non seulement au temps de travail, mais aussi à l'amélioration des conditions Ce furent d'abord les 40 heures, grâce au Front populaire, puis les 39 heures, en 1982, enfin les 35 heures obligatoires dans toutes les entreprises, à partir de 2002. À l'orée d'une élection présidentielle, je tiens à saluer nos collègues du groupe CRCE pour avoir mis ce débat à l'ordre du jour. Ce sujet mérite selon moi d'être abordé sereinement et sérieusement, loin des clichés nous expliquant que les Français sont plus enclins à favoriser leurs loisirs, qu'ils ne travaillent pas suffisamment en comparaison de leurs homologues européens, loin aussi de l'idée qu'il suffirait d'être volontaire, tout simplement, pour trouver du travail. « Le partage du temps de travail, un outil pour le plein emploi ? » : la question est de savoir s'il faut travailler moins pour travailler tous. On pourrait répondre assez aisément que les 35 heures n'ont pas permis de résorber le chômage de masse et que les exonérations concédées à l'époque n'ont pas eu les retombées espérées. On pourrait également se dire qu'une meilleure répartition du travail permettrait une meilleure répartition des richesses, mais tel ne fut pas le cas en 2002. Dans un contexte de flambée des prix de l'essence, du gaz et de l'électricité, les Français sont-ils prêts à travailler moins pour gagner moins ? Je ne le pense pas. L'idée n'est pas de remettre en cause les 35 heures, qui sont un acquis social, mais simplement d'en dresser un constat lucide : si elles ont permis davantage de temps libre, leur effet sur l'emploi et la réduction du chômage fut très limité. Le prisme de la réduction du temps de travail, s'il n'est pas à éliminer, me paraît insuffisant pour réduire le chômage.

Il n'est plus possible de se satisfaire d'une France où le taux de chômage des jeunes avoisine les 20 % et où, en même temps, des commerces ferment, des boulangers et des bouchers recherchent désespérément des apprentis, des emplois restent non pourvus. pourvus. Oui, il s'agit souvent de métiers difficiles, aux horaires décalés, mais il faut peut-être informer davantage et mieux communiquer sur ces professions de grande qualité. Un débat sur le travail nous oblige également à réfléchir à ce que celui-ci apporte en fait de relations sociales et d'estime de soi, au-delà de la rémunération. À cet égard, le combat contre le chômage de longue durée mérite d'être mené tant ledit chômage peut avoir des effets dévastateurs pour les principaux concernés. L'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », conduite depuis 2016, permet notamment de ramener vers l'emploi les publics qui en sont le plus éloignés, des jeunes, des femmes et des personnes peu diplômées. Si la crise sanitaire que nous connaissons a perturbé certaines expérimentations, il faut continuer à encourager ces projets qui sont de vrais outils d'insertion sociale. Le travail doit certes être encouragé : il reste le meilleur moyen de sortir de la précarité. Mais il nous faut également être pragmatiques.

Dire tout cela ne sert à rien si l'on ne prend pas en compte l'évolution du travail ces dernières années. Au premier rang de ces transformations, le télétravail est venu bouleverser les habitudes durant le confinement. Au-delà même du nombre d'heures de travail, on observe un changement de paradigme : émerge une approche davantage centrée sur le nombre de jours de travail. Certains pays mettent en place la semaine de

Plus largement, un débat sur le travail mériterait également que l'on s'interroge sur la place du salarié dans l'entreprise la revalorisation de l'intéressement et la hausse de sa participation au sein des conseils d'administration des entreprises.

Pour elles, cela signifie une fragilité financière, un sentiment d'inutilité et de relégation sociales ou, à tout le moins, une difficulté à concilier projet personnel et utilité sociale. Le débat qui nous réunit aujourd'hui autour du partage du travail n'est pas nouveau, il est indissociable de l'évolution des conditions de travail et de l'organisation du travail tout au long de la vie. Depuis 1919, des lois résultant de plusieurs décennies de lutte et de revendications syndicales ont scandé un mouvement historique de réduction du temps de travail au cours du XX siècle. Ces réformes promues par des gouvernements de gauche ont permis de réduire le temps de travail et de repenser la relation au travail. Je citerai les 39 heures et la cinquième semaine de congés payés instaurées après l'élection de François Mitterrand en 1981, ainsi que les deux lois de 1998 et 2000

Ces allègements de la durée du travail ont aussi permis un meilleur équilibre entre le travail et le temps personnel et familial. Cette dynamique de progrès et de partage du travail est freinée depuis vingt ans et, surtout, les inégalités se sont accrues entre les travailleurs. La baisse du temps de travail la plus importante est due, pour un quart, au développement du temps partiel, le plus souvent subi, le plus souvent par des femmes, qui exercent des métiers imposant des temps réduits ou doivent s'occuper de leur famille. Depuis 2003, les salariés à temps complet ont vu leur temps de travail augmenter. Le Président de la République a affirmé, lors de la présentation de son plan d'investissement France 2030, que « notre pays travaille moins que les autres ». Les chiffres démentent

et cause de nouvelles formes de souffrance au travail ; ainsi le nombre de burn-out a-t-il explosé. La crise du covid a poussé de nombreux salariés à s'interroger sur la place que devait occuper le travail dans leur vie. Ceux-ci aspirent à organiser leur vie professionnelle de manière plus libre, alors qu'ils sont plus nombreux à travailler de manière autonome et à distance. Les jeunes générations aiment le travail, y compris les travaux pénibles, mais souhaitent des compensations à la pénibilité et aux contraintes horaires- je pense par exemple au secteur de la restauration. Notre société doit s'adapter à un monde qui devient moins créateur d'emplois et transforme notre rapport à l'existence, au travail, à la protection sociale ou, tout simplement, à la préservation de notre santé et de notre bien-être. d'un choix de société ambitieux ; c'est par davantage de solidarité que le travail retrouvera sa véritable valeur, redonnant du sens à nos métiers et compensant les pénibilités. Plusieurs pays ont suivi notre exemple de réduction du temps de travail. Notre voisin espagnol a décidé de lancer une expérimentation. En 2022, ce sont 200 entreprises volontaires qui testeront la semaine de quatre jours sans baisse de salaire. La durée du travail considérée tout au long de la vie fait débat en France. La réforme des retraites préconisée par Macron et par d'autres à droite prévoit un recul de l'âge de la retraite. Un retour en arrière a déjà eu lieu en 2017 la suppression de plusieurs critères de pénibilité ouvrant droit à compensations : port de charges lourdes, vibrations, postures postures douloureuses, présence d'agents chimiques dangereux. Près de 300 000 personnes ou emplois potentiels, ces derniers principalement pourvus par des ouvriers dont les conditions de travail sont pénibles, se retrouvent

Avec les partenaires sociaux, le Gouvernement pourrait se saisir du sujet de l'organisation du temps de travail tout au long de la vie en y incluant la question des retraites, afin d'aboutir à un accord national interprofessionnel et à une négociation par branche. Une réduction du temps de travail intégrant les critères de pénibilité serait une réponse au problème du chômage structurel dans notre pays, une manière d'éviter les fins de carrière anticipées dues à des inaptitudes au travail et d'améliorer le bien-être au travail pour tous. La

il s'agit de réduire le temps de travail pour permettre aux salariés de profiter davantage de leur vie familiale, sociale, culturelle, sportive et démocratique. Troisièmement, il s'agit de mieux répartir les richesses pour participer à l'amélioration des conditions de travail, des salaires et de vie des salariés. Ces idées sont louables ... Pour autant, la crise que nous vivons nous apporte à ce sujet de multiples enseignements. Alors que les conjectures laissaient imaginer en 2021 la destruction de plus de 230 000 emplois et tandis que la pandémie continue à perturber fortement le marché du travail, la réalité est bien différente. Le chômage baisse et atteint les 8 %, soit son niveau le plus bas depuis quinze ans. Le taux d'emploi est en hausse, à près de 66 %. Selon la Dares, le nombre d'emplois vacants a augmenté très fortement, de +33 %, par rapport à la situation d'avant crise et de façon généralisée dans tous les secteurs. Les embauches en CDI, 416 000 comptabilisées en novembre 2021, n'ont jamais été aussi hautes depuis 2006. Ces chiffres, parmi bien d'autres, laissent présager que le plein emploi est à notre portée, à tout le moins que la trajectoire n'a jamais été aussi positive depuis plus de trente Ces résultats ne sont en rien le fruit du hasard. Ils sont liés à des choix politiques forts, dont nombre concernent l'organisation du travail. Je citerai quelques exemples. Tout d'abord, je citerai la réforme du droit du travail, qui a laissé une bien plus grande place aux négociations au sein des entreprises ou des branches, l'aménagement plus souple de l'organisation du travail, en particulier grâce au développement du télétravail. Il faut noter, ensuite, la volonté affichée de favoriser l'entrée des jeunes sur le marché. Je pense au plan « 1 jeune, 1 solution » et à l'apprentissage. le plan d'investissement dans les compétences et la mobilisation de 15 milliards d'euros, lancé en 2018, qui a eu pour objectif, à travers la formation, d'insérer durablement dans l'emploi les demandeurs d'emploi, notamment les jeunes. Aujourd'hui, plus de 1 million de personnes en recherche d'emploi sont ainsi formées chaque année, contre 600 000 personnes avant ce plan. une réforme forte et assumée de l'assurance chômage, avec deux lignes principales : faire que la rémunération soit plus importante au travail qu'au chômage, et pousser les entreprises à sortir de la logique des CDD de très court terme. C'est bien cet ensemble de mesures qui a entraîné la création d'emplois et qui nous a permis d'éviter une crise sociale de grande ampleur. Au-delà de l'organisation du travail, un deuxième élément, peut-être le plus essentiel, est la réforme de la formation continue. En 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a levé les discriminations persistantes dans notre pays et donné les a levé les discriminations persistantes dans notre pays et donné les moyens de créer cet espace d'émancipation qui permet aujourd'hui à nos concitoyens de choisir librement leur parcours, en bénéficiant de protections collectives. personnel de formation (CPF), avec en 2021 plus de 2 millions de personnes inscrites à une formation, contre 630 000 en 2019, en est une preuve incontournable. Les Français sont désormais libres de se réorienter, de changer de spécialité pour être en adéquation avec le marché du travail et avec leur ambition personnelle. L'épanouissement au travail n'est plus une utopie. Trouver du sens dans ce que l'on fait, travailler sur des projets impactants ou relever des challenges au quotidien, partager des valeurs communes ou être reconnu par ses pairs et sa hiérarchie sont autant de facteurs d'épanouissement et d'émancipation. C'est ainsi que se construit une meilleure concordance entre les besoins des entreprises et les choix assumés de ceux qui se forment. En résumé, donner plus de souplesse aux entreprises, libérer les énergies des salariés, en ayant confiance dans leur capacité à se former et pousser à la négociation de terrain sont les plus forts atouts pour faire baisser le chômage et créer de la richesse.

simplement parce que ce temps libéré n'a pas été créateur d'une rémunération plus importante. Elle a en revanche eu pour conséquence la multiplication du recours aux emplois précaires, parfois non déclarés, pour arrondir les fins de mois. Elle a, de plus, engendré des tensions préjudiciables envers les salariés dans les petites entreprises. Supprimer quatre heures de travail par semaine et par salarié dans une petite structure ne construit pas un temps plein. Le corollaire de cette réforme est la création d'heures supplémentaires dans le meilleur des cas. Elle s'accompagne d'une obligation de productivité accrue la plupart du temps. Être stressé, car débordé, ne participe en rien à l'épanouissement. En partant d'une intention louable, mais idéologique, on obtient malheureusement le résultat inverse. Enfin, et c'est aussi l'intérêt de ce genre de débat, qu'il me soit permis de sortir un peu du cadre contraignant qui consiste à réfléchir en termes de « plus ou moins d'heures travaillées ». Il pourrait être utile de se rappeler que les femmes et les hommes ne sont pas des machines. Vouloir toujours résumer le travail à un décompte du temps passé au travail est terriblement réducteur. Ainsi, en fonction de sa forme et de ses soucis, un salarié peut un jour accomplir une tâche en une heure, et en deux heures un autre jour. J'ai la conviction, l'ayant moi-même mise en place par la voie de la négociation, que cette piste, si elle est partagée et bien comprise, est facteur d'épanouissement pour les salariés, qui organisent ainsi beaucoup mieux leur temps de travail, et créateur de richesse pour l'entreprise. Sur un tel sujet, notre rôle est également de sortir de la binarité quasi idéologique du décompte du temps de travail, mais aussi d'intégrer tous les facteurs possibles d'épanouissement et de réussite partagés entre les salariés et les entreprises. Ce gouvernement en a fait la démonstration par toutes ses réformes, mais il reste encore de nombreuses pistes à explorer ! La parole

L'instauration de l'euro nous a permis, malgré les déficits, de ne pas dévaluer notre monnaie, d'où notre facilité à vivre avec des déficits. Depuis vingt ans, nous n'avons pas su prendre les mesures pour rétablir l'équilibre budgétaire. En 1983, au temps du franc, Jacques Delors, au sein du gouvernement d'union de la gauche, avait été contraint, pour ne pas trop dévaluer la monnaie, à prendre des mesures d'austérité alors acceptées par les partis de gouvernement. En 1998, le commerce extérieur français était excédentaire alors que l'Allemagne affichait un déficit commercial. En 2020, les situations sont inversées. Que s'est-il passé ?

cette part du PIB est passée de 18 % à 26 %, avec des emplois à la clé. Pourquoi une telle évolution ? J'y vois trois raisons principales. Première raison : l'évolution des coûts de production pour les entreprises. En Allemagne, le chancelier Schröder, avec le soutien des syndicats, a gagné l'entrée dans l'euro grâce aux rigueurs des années 2000. Au même moment, nous nous autorisions une baisse du temps de travail, aggravant l'augmentation du coût du travail, et donc réduisant la compétitivité des entreprises, malgré les aides publiques mises publiques mises en place pour accompagner le passage aux 35 heures. Deuxième raison : l'euro a stimulé le commerce intra-européen en facilitant les transactions, ce qui a renforcé la nécessaire compétitivité entre les entreprises. Toute différence de prix, même faible, a une importance capitale. Les emplois industriels se sont concentrés dans les zones les plus productives. Troisième raison : dans une économie de marché

pas d'Europe sociale, dotée d'un salaire minimum homogène dans toute la zone. D'où la délocalisation des industries vers les pays de l'Est. a été cité, je pourrai également parler de la Corrèze et de BorgWarner. Pourtant nous devons absolument réindustrialiser notre pays pour financer une protection sociale indispensable : sécurité sociale, assurance chômage, retraites, aides sociales,

Tel est le chemin d'une véritable Europe sociale vers laquelle nous devons nous engager. Il serait souhaitable de parler de la répartition des richesses dans notre pays. Mais cette meilleure répartition ne doit pas être nécessairement synonyme de davantage d'impôts. Le plus important est d'abord de créer des richesses avant de les répartir. Ensuite seulement il sera possible d'augmenter les salaires,

Pour créer de l'emploi et des richesses, il faut plus d'entreprises compétitives par rapport à nos concurrents européens. Votre proposition, généreuse dans son principe, de réduire le temps

mes chers collègues, je remercie mes collègues du groupe CRCE d'avoir mis à l'ordre du jour, dans ce contexte de crise sanitaire qui se prolonge, ce débat sur le thème « le partage du travail : un outil pour le plein emploi Au fond, ce sujet est d'actualité puisque le marché du travail a été plus que jamais à l'épreuve de la crise sanitaire depuis 2020. Le sujet est revenu sur le devant de la scène à l'occasion de la Convention citoyenne pour le climat, laquelle a proposé une réduction du temps de travail à 28 heures-

un peu plus, la création de croissance supplémentaire ». Comment faire pour relancer une économie qui se déconfine ? Faut-il travailler plus, produire plus, pour rattraper le temps perdu ? Faut-il, au contraire, partager le temps de travail entre tous, avec ou sans baisse de rémunération, pour lutter contre le chômage ?

Les pays qui ont le taux de chômage le plus bas sont donc quasiment au plein emploi : l'Allemagne est à 3,3 %, le Royaume-Uni à 4,2 %, les Pays-Bas à 2,7 % ; la Norvège et la Pologne présentent un taux respectif de 3,6 % et de 3,4 et de 3,4 %., selon l'enquête sur les forces de travail conduite par Eurostat dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, en France, la durée effective annuelle moyenne du travail était en 2019 de 1 680 heures pour les salariés à temps complet- vous avez eu raison, monsieur le secrétaire d'État, de le souligner -, soit le plus faible taux des pays de l'Union européenne après la Suède.

Sans en tirer d'autres conclusions, nous pouvons considérer que les pays connaissant le plein emploi au niveau européen sont largement ceux dans lesquels le temps de travail est supérieur au nôtre. Le deuxième point consiste à observer les suites du passage de 39 heures à 35 heures prévu par les lois Aubry I et II.

comme Nicolas Bouzou, économiste libéral et directeur du cabinet Asterès, estiment que ce sont les mesures d'accompagnement et d'allégement de charges qui ont créé des emplois, mais que les 35 heures en elles-mêmes n'ont pas eu d'impact positif avéré sur l'emploi. état de cause, tous concluent que les 35 heures ont dégradé les finances publiques, car les baisses de cotisations n'ont pas été financées par le surplus de croissance attendu. Très bien ! Par ailleurs, l'Institut Montaigne estime qu'un retour aux 39 heures permettrait d'économiser 7 milliards d'euros par an

Le troisième point concerne l'impact d'une baisse du travail sur le secteur public. Il est en effet fondamental, pour des raisons évidentes d'équité, d'associer le secteur public au secteur privé pour conduire cette réflexion. Or, si l'on revient sur les 35 heures, plusieurs travaux ont été conduits, dont ceux de notre collègue Albéric de Montgolfier : il chiffrait à 21 milliards d'euros, sur la période 2005-2015, le coût du passage aux 35 heures pour les seules fonctions publiques d'État et hospitalière, du fait de l'embauche de 50 000 agents supplémentaires. Il s'agit donc, si l'on aborde la question de la baisse du temps de travail dans la fonction publique, d'envisager l'équilibre financier et notre capacité à financer une telle réforme, à l'heure où la Cour des comptes souligne que « l'impact sur les finances publiques de la crise sanitaire et des mesures prises pour y faire face est considérable » et que « la soutenabilité des finances publiques s'inscrit dans le temps long avec des manifestations de perte de confiance qui peuvent être rapides et brutales » ... Dernier point : parce que la logique du temps de travail répond avant tout à une productivité et que celle-ci est différenciée, avec des secteurs économiques en surcharge de travail et d'autres au contraire en sous-charge, nous ne pouvons que nous réjouir que les 35 heures n'aient en réalité duré que de 1998 à 2002. Le monde bouge, évolue et emporte avec lui un flot permanent de mutations en tous genres, dont la digitalisation de l'économie, la plateformisation, le télétravail et bien d'autres phénomènes. Ce qu'il reste des 35 heures, c'est un cadre rigide et un management d'outre-tombe, alors qu'il faudrait être plus flexible et valoriser davantage l'intelligence. Félicitions-nous donc que les 35 heures aient progressivement évolué des baisses de cotisations plus larges et une augmentation du contingent d'heures supplémentaires. Nos entreprises ont ainsi pu s'adapter à un marché concurrentiel et changeant, tout en créant des emplois. Pour ma part, je pense que plus on travaille, plus il y a de travail.

Laissons à nos entreprises, sur la base d'un cadre flexible et souple, la possibilité de s'adapter. Il y va de la pérennité de leur performance et parfois même de leur survie. et par des réorganisations de modèle managérial en profondeur, que nous gagnerons le pari de l'emploi et de l'appétence de chaque collaborateur pour son poste et son activité. Eu égard à la logique d'équilibre des comptes sociaux et de leur pérennité, chacun a bien compris que que l'équation était assez simple : à défaut de réformer nos systèmes de retraite en allongeant notre temps de travail, nous appauvrirons les retraités et nous creuserons les déficits. La campagne électorale à venir permettra à chacun de faire des choix éclairés et notre groupe politique fera, comme tel a toujours été le cas, le choix de la responsabilité, de l'analyse objective et du courage politique, dans une perspective de plein emploi et d'équilibre des comptes sociaux ! Excellent

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le partage du travail est un outil pour le plein emploi, et je remercie le groupe CRCE d'avoir posé ce débat dans notre hémicycle. Au-delà, c'est aussi un outil de la transition écologique pour le plein emploi, pour retrouver le sens du travail, pour la santé des travailleurs, pour le partage des richesses, pour une société heureuse produisant selon nos besoins et non pour le profit de quelques-uns.

celle des hommes cadres est de 84 ans, soit 6,4 années de plus. C'est ainsi la double peine pour les ouvriers : ils vivent moins longtemps pour profiter de leur retraite et développent, à cause d'un travail harassant qu'ils occupent trop longtemps, davantage de handicaps et d'incapacités physiques liés à la pénibilité du travail. Cette injustice est insupportable. Oui, le partage du travail est un outil majeur de la transition écologique, dans la justice sociale, parce qu'il permet une désintensification du travail, protectrice pour la santé des travailleurs, une meilleure qualité de vie et du temps libéré pour les liens sociaux, et parce qu'il permet de prendre en compte, d'anticiper et d'accompagner l'inexorable et heureuse diminution du travail humain dans certaines branches, liée à la robotisation, et son transfert dans d'autres. Ce mouvement de réduction du temps de travail doit se faire de différentes manières. Fini le temps des directives strictes venues d'en haut, s'appliquant de manière uniforme, sans prise en compte des réalités du travail mouvement doit se faire au profit des salariés. Toutes les possibilités doivent être mobilisées pour le partage du travail et la réduction du temps de travail : à l'échelle de la semaine, de l'année, avec les congés payés ; ou à l'échelle de la vie, avec l'abaissement de l'âge de départ à la retraite et des années libérées pour des projets de professionnalisation et de formation. Le travail se transforme et nécessite moins de main-d'oeuvre, pour une production égale, voire supérieure. Alors que les progrès constants de la technologie, de notre système éducatif, de nos infrastructures publiques ont permis aux entreprises de produire davantage de richesse avec autant de salariés, la réduction du temps de travail est une manière de faire bénéficier les travailleurs de ces gains ainsi qu'un outil plus juste au service du partage équitable du travail entre tous et toutes. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, la machine s'est enrayée. Les gains de productivité auraient-ils arrêté de croître ? Absolument pas ! La productivité horaire des Français est l'une des plus importantes au monde, cela a été Le temps de travail effectif tend à augmenter avec les assouplissements récents, les salaires stagnent, voire diminuent avec la pression du chômage et l'explosion de l'ubérisation. Il a été absorbé par les entreprises dans l'illusoire « travailler plus pour gagner plus » qu'aucun gouvernement gouvernement n'a été capable de remettre en cause. Qui peut encore y croire à l'heure où le travail est plus mal partagé que jamais, et que certains, qui frôlent quotidiennement le burn-out, côtoient des intermittents de l'emploi précaire- en augmentation -, peinant à aligner quelques heures de missions par semaine pour remplir le frigo Le « travailler plus pour gagner plus » est terminé, autant que la course folle au tout-productivisme. Le sacrifice des travailleurs qu'on presse comme des éponges sur l'autel de la croissance ne peut plus durer

Permettons aux Français de retrouver la maîtrise de leur vie, de s'investir dans la vie citoyenne, dans la vie associative ou de prendre davantage de temps pour leur émancipation personnelle ! Permettons aux Françaises et aux Français qui ont commencé à travailler jeunes et à ceux qui occupent des métiers difficiles de partir à la retraite plus tôt et de profiter d'un temps de repos mérité. Pour cela, prenons vraiment en compte les critères de pénibilité dans le calcul de la retraite : à la place d'un système hyperindividualisé où l'on peine à accéder à ses droits, prévoyons un système de garanties collectives fortes ! Mes chers collègues, il est l'heure

un vecteur de l'égalité entre les femmes et les hommes. La réduction de quelques heures par semaine de la durée légale de travail pour un temps plein afin d'offrir une meilleure qualité de travail, sans perte de salaire, correspond à une aspiration de plus en plus forte dans notre société. La sociologue Dominique Méda, autrice de nombreux ouvrages sur le travail et les politiques sociales, a parfaitement analysé ce sujet et rappelé que l'enjeu de la réduction du temps de travail

augmentaient : « Le temps est source d'inégalité massive entre les femmes et les hommes. » Le partage du temps domestique et familial entre les femmes et les hommes est indispensable pour éviter qu'il ne repose exclusivement sur les femmes. Lors du passage aux 35 heures, l'Institut national d'études démographiques (INED) a mesuré que le temps moyen consacré aux tâches domestiques avait augmenté de douze minutes par jour chez les hommes. Si ce progrès demeure très relatif, notamment en matière de charge mentale, qui repose encore en majorité sur les femmes, la baisse du temps de travail participe toutefois à l'amélioration du partage des tâches entre les sexes. Mais réduire le temps de travail à 32 heures hebdomadaires aurait également une incidence sur les temps partiels imposés, en permettant à de nombreuses femmes d'accéder à un temps plein. Selon l'Insee, la différence de temps de travail est la première cause des 28 % d'écart salarial entre hommes et femmes. écart se répercute sur la retraite et explique l'essentiel des 40 % d'écart de pension entre les hommes et les femmes. De plus, il n'est pas inutile de rappeler ici que les temps partiels imposés et les politiques d'exonération de cotisations sociales

Les opposants à la réduction du temps de travail sont souvent les partisans des contrats courts et des temps partiels. Les mini-jobs et autres contrats courts sont pourtant autant d'emplois précaires qui renforcent les inégalités entre les femmes et les hommes. Enfin, la réduction du temps de travail doit s'accompagner d'un renforcement des moyens d'intervention des salariés dans les entreprises. Cela passe par le rétablissement des CHSCT (comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et par de nouveaux droits d'intervention, comme le droit de veto des salariés. La réduction du temps de travail à 32 heures n'est pas une lubie des organisations syndicales et de certains partis politiques, dont le nôtre. Elle constitue la réalité dans certaines entreprises françaises, comme Bosch à Vénissieux, Welcome to the Jungle ou Love Radius dans le Var. En Espagne, depuis le mois de mars 2021, le gouvernement a décidé d'engager une expérimentation de la semaine de 32 heures sur quatre jours avec maintien des salaires. Cette expérience porte sur 200 entreprises et plusieurs milliers de salariés. Enfin, le mouvement « 4 Day Week » mène campagne en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Irlande en faveur d'une réduction du temps de travail. En conclusion, la réduction du temps de travail est un projet politique global qui repense la place de l'individu dans l'entreprise et la cité. la cité. Elle vise à l'amélioration des conditions de vie en permettant, notamment, de mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, et de disposer de temps pour soi, pour les autres, pour les loisirs, la culture ou pour des engagements associatifs par exemple. Un passage à quatre jours par semaine aurait également un rôle positif sur la santé des salariés. Ce serait aussi un outil de réduction des déplacements, ce qui ne peut être que bénéfique pour l'environnement et l'amélioration des conditions de travail, et un levier pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Contrairement à ce qu'a dit le Président de la République, la France n'est pas le pays où l'on travaille le moins en Europe, ainsi que l'a montré ma collègue Cathy Apourceau-Poly. Au contraire, nous avons une durée moyenne hebdomadaire parmi les plus élevées, ainsi qu'une productivité de vingt points supérieure à la moyenne européenne. Cette productivité doit être partagée pour permettre le travail de toutes et tous, des femmes et des hommes, des jeunes comme des anciens. Alors, en 2022, engageons-nous dans cette voie de progrès social ! La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens à remercier le groupe CRCE pour le débat qu'il propose. La question du partage du temps de travail comme levier pour atteindre le plein emploi à la fin du quinquennat implique d'abord de faire le bilan de l'action du Gouvernement. La politique de l'emploi en France est un échec total. Le chômage se stabilise dans notre pays, mais à un niveau trop élevé, auquel nous avons trop tendance à nous habituer. Je présume que le Gouvernement vantera les bons chiffres d'un taux de chômage se stabilisant à 8 %, c'est-à-dire « mieux qu'avant la crise ». C'est exact, mais c'est encore insuffisant

Pourtant, depuis quarante ans, tous les outils ont été mis sur la table. François Mitterrand disait en 1993 : « Contre le chômage, on a tout essayé. » D'autres répondaient : « Sauf ce qui marche ! y compris le partage du travail avec les 35 heures de Mme Aubry, qui n'ont pas été la solution pour tendre vers le plein emploi. Peut-être certains ici diront-ils que les 32 heures permettront de faire face à la robotisation, à internet et à la raréfaction de l'emploi. Nous n'y croyons pas : les 32 heures n'auront pas davantage d'effet que les 35 heures. Certains grands économistes annoncent que l'automatisation implique une réduction de l'emploi et, par conséquent, une nouvelle répartition du temps de travail. Pour ma part, j'estime que le partage du travail n'est pas le premier outil pour tendre vers le plein emploi. En effet, lorsqu'une société a un niveau de chômage structurel se situant aux alentours de 9 % à 10 %, elle est dans une phase de son existence

L'état de récession et les crises laissent des séquelles que la répartition du temps de travail ne résout pas. La désindustrialisation et la tertiarisation désindustrialisation et la tertiarisation de notre économie maintiennent le chômage dans un lit douillet et les chômeurs dans l'enfer des oubliés. Le constat est là. En s'accommodant trop longtemps de 10 % de chômage structurel, la France est touchée par une apathie économique et sociale : des générations, des familles entières qui vivent dans le chômage, avec pour corollaire la désagrégation du statut social et de l'estime de soi. Monsieur le secrétaire d'État, j'aimerais connaître vos propositions sur les moyens de lutter à l'avenir contre l'inadéquation que nous observons aujourd'hui entre secteurs recruteurs ne trouvant pas d'employés et secteurs saturés.

d'anticiper la France de 2040. Il faut désengorger le tertiaire au profit des nouvelles industries. Il faut également acter la décentralisation économique vers nos territoires, protéger nos brevets et éviter la fuite à l'étranger des personnes hautement qualifiées. Il sera également nécessaire de mener une réflexion sur le travail lui-même.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, confinements et vagues épidémiques successives nous ont incités en 2020 à nous interroger sur la vie d'après. Le travail, notamment son organisation, n'y a pas échappé. Aujourd'hui, que reste-t-il de ces envies d'autrement ? Quand philosophie, sociologie et autres sciences humaines envisagent le travail sous des angles parfois totalement différents, l'approche économique confond souvent emploi et travail. et travail. Ainsi partager le travail nous permettrait-il de trouver le plein emploi. L'équation est tentante, mais l'approche arithmétique ne suffit pas. Qu'est-ce que le plein emploi ? Doit-on le vouloir à tout prix et, surtout, à quel prix ? Peut-on le considérer comme désirable quand il se compose pour partie de salariés dont le temps de travail partiel est subi, quand il n'atteint même pas les 24 heures hebdomadaires ? Posons-nous la question. Quand ce travail est précaire, partiel, pénible- parfois même il cumule ces trois caractéristiques -pour certains, plutôt devrais-je dire « certaines » puisque majoritairement ce sont des femmes qui occupent ces postes, est-ce enviable, est-ce souhaitable ? Là aussi, interrogeons-nous. Un travail à la mesure de chacune et de chacun est possible. C'est l'une des approches des territoires engagés dans la démarche des « territoires zéro chômeur de longue durée Dans mon département, en Loire-Atlantique, c'est l'objectif que s'est fixé le territoire de Pont-Château, dont les efforts ont permis d'aboutir à la labellisation « territoire zéro chômeur de longue durée » à la fin de l'année dernière. Partant du constat selon lequel personne n'est inemployable et qu'une personne privée d'emploi coûte plus à la société qu'une personne salariée,

Ces dernières interviennent dans des secteurs où l'offre de services n'est localement assurée par aucun acteur économique public ou privé. À Pont-Château, c'est dans le domaine de la réutilisation de bois et d'offres de services à la personne qu'interviendront les salariés à durée indéterminée nouvellement embauchés, après avoir été durablement privés d'emploi du fait soit de handicap, soit d'accident de la vie. D'autres territoires enclenchent la démarche. Dans mon département toujours, la commune de Loireauxence a elle aussi décidé de se mobiliser. Le pays d'Ancenis, en Loire-Atlantique, est reconnu pour détenir un taux d'emploi record. On y atteint même le plein emploi dans la ville-centre. Or la situation est un trompe-l'oeil : il y persiste un chômage résiduel. Les causes en sont multiples : difficultés de mobilité, absence d'offres en adéquation avec les compétences mobilisables et disponibles, souhait des personnes de sortir durablement de la précarité instaurée par de de petits contrats saisonniers ou des missions de courte durée, ou enfin des situations personnelles imposant de trouver un emploi répondant aux obligations familiales- et je pense là aux femmes seules avec enfants. Derrière les chiffres, il y a des réalités d'hommes et de femmes.

est vrai que nous posons la question du partage de la valeur ajoutée. Oui, nous devons augmenter la taille du gâteau ; je rappelle toutefois que près de 6 millions de nos concitoyens sont sans emploi, et n'ont donc aucune part de ce gâteau ... À l'inverse, les actionnaires et les dirigeants des grandes entreprises se réservent la meilleure part. Nous

Je rappelle en outre que, durant la crise sanitaire, 200 000 personnes ont été radiées des listes pour rejoindre le halo du chômage. Comme l'indiquait notre collègue du groupe RDSE, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un taux de chômage des jeunes à 20 %. Je note les points d'accord avec les groupes socialiste et écologiste sur la nécessité de réduire le temps de travail, et je partage les propos de Marc Laménie concernant les difficultés des territoires sinistrés. réduire le temps de travail, nous devons aussi aux travailleurs à temps partiel, qui sont souvent des travailleuses, d'augmenter leur temps de travail. La bataille pour le temps libre a toujours été un combat. Aujourd'hui encore, le temps disponible demeure le reflet des inégalités.

contre 40,4 heures pour les pays de l'OCDE. Nous sommes donc pleinement dans la moyenne européenne, et non en dehors ! Contrairement à nos collègues de droite, nous considérons qu'en allongeant la durée de cotisation et en repoussant l'âge de départ à la retraite, on maintient des salariés en activité alors que leurs emplois pourraient être occupés par des jeunes

En posant la question de la diminution du temps de travail, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste s'inscrit dans un projet de transformation de la société où le fruit des richesses créées profiterait en priorité au plus grand nombre, et notamment à celles et à ceux qui les produisent par leur travail. Une meilleure répartition du travail permettrait à toutes et tous de travailler dans de meilleures conditions, de préserver l'environnement- cela a été dit à plusieurs reprises -, d'aller dans le sens de l'égalité femmes-hommes et de mieux rémunérer le travail en augmentant les salaires,

je vous remercie